La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 1 juin 2023 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, alimentaire. Madame la ministre, ma question porte sur l'impact financier des mesures de prévention de la prédation, qui ne sont pas sans conséquence sur l'équilibre économique des exploitations d'élevage. Face à l'inquiétante prolifération du loup, les éleveurs sont contraints de renforcer les moyens de protection dont ils assurent le cofinancement au minimum à hauteur de 20 %. Ils sont souvent amenés à faire une avance de trésorerie qui, dans le meilleur des cas, leur sera remboursée un an plus tard. Toutes ces mesures de protection ont un coût pour des éleveurs de plus en plus découragés au point d'envisager l'arrêt de leur activité. À quelques mois de l'entrée en vigueur du prochain plan national loup, sur lequel les arbitrages seront rendus en juillet êtes-vous favorable à une prise en charge intégrale des équipements de protection, au vu du nombre de victimes ? Accepteriez-vous d'autoriser le remplacement des animaux tués plutôt que d'indemniser les éleveurs qui en feraient la demande, et ce afin d'éviter d'alourdir la fiscalité des exploitations ? Enfin, seriez-vous prête à examiner la demande des éleveurs de pouvoir déduire

pour qu'ils mettent en oeuvre des mesures de protection des troupeaux : aide au gardiennage par les bergers, achat de clôtures, achat et entretien de chiens de protection, accompagnement technique. Un dispositif d'accompagnement technique des éleveurs a été lancé en 2018 pour optimiser l'efficacité des moyens de protection.

En novembre 2021, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, M. Joël Giraud, a annoncé le déblocage d'une somme de 24 millions d'euros sur les 16 milliards d'euros du Ségur de la santé, afin d'aider à la réhabilitation complète du du service, affirmant ainsi sa volonté que les petits hôpitaux du territoire ne soient pas oubliés. Ce projet de rénovation avait obtenu le feu vert de l'agence régionale de santé (ARS) en septembre 2018. En effet, l'établissement morlaisien n'est pas un simple hôpital de proximité : il s'agit aussi d'un hôpital de recours territorial offrant de nombreuses spécialités, médecine interne ou la neurologie, et un volet de recherche et développement très intéressant pour les jeunes médecins. L'aide indispensable que représente cette enveloppe de 24 millions d'euros de l'État reste cependant insuffisante au vu du coût du chantier. En effet, la réhabilitation du pôle MCO, devenu vétuste, implique un investissement de 94 millions d'euros, qui doit permettre de s'adapter à la nouvelle offre de soins. Ce budget, initialement fixé à 80 millions d'euros, a dû être réévalué en raison de la hausse du coût des matières premières.

L'assiette financière globale du projet a peu varié depuis son origine, dans la mesure où la direction de l'établissement est parvenue à limiter les conséquences de la hausse du coût des matières premières grâce à des révisions itératives du projet, notamment en mettant l'accent sur la restructuration du bâtiment existant et en minorant les surfaces à construire.

L'ARS et le ministère demeurent attentifs au projet d'investissement du CHPM. Celui-ci s'inscrit pleinement dans les orientations du Ségur de la santé qui, je le rappelle, dans son volet investissement tout à fait inédit de 19 milliards d'euros, a permis d'engager et de soutenir la réhabilitation et la reconstruction de très nombreux établissements de proximité à travers le territoire.

porte sur le maintien d'une offre de soins hospitaliers sur le territoire de Saint-Louis dans le Haut-Rhin. Dimanche dernier, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur ce territoire en soutien à leur hôpital. En effet, à la suite de la fermeture de la clinique des Trois-Frontières et de la reprise de son activité par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), beaucoup craignent que le maintien dans l'agglomération d'une offre de soins de qualité, adaptée aux besoins de leur territoire et de ses plus de 80 000 habitants, ne soit pas assuré. Le GHRMSA peine à mettre en place le projet prévu

Madame la ministre, quelles sont vos intentions à ce sujet et quels moyens entendez-vous mettre en place pour faire face à cette situation préoccupante ? Afin de rétablir le lien de confiance entre les parties prenantes, êtes-vous prête à envisager un comité de pilotage ?

La reprise à 100 % de l'hôpital de Saint-Louis- ancienne clinique des Trois-Frontières -par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) est le résultat d'une procédure de redressement judiciaire qui a permis de garantir la continuité de l'activité. Elle est le gage de la durabilité du site. L'hôpital de Saint-Louis vient d'être labellisé « hôpital de proximité » par l'ARS, ce qui contribue à sécuriser ses financements à moyen terme. De nombreux efforts ont été consentis pour assurer la pérennité du site et l'offre de consultations

Malgré une démographie médicale difficile, le GHRMSA a pour objectif d'augmenter le nombre de lits et de places du service de médecine et des SSR, de développer de nouvelles consultations avancées spécialisées en chirurgie, en rééducation, en diabétologie et en neurologie, de déménager les activités de psychiatrie sur le site de l'hôpital et de créer un hôpital psychiatrique

De manière générale, si 87 % des territoires métropolitains sont considérés comme des déserts médicaux, la situation est plus prégnante encore dans les territoires transfrontaliers où toujours plus de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants franchissent chaque jour la frontière pour travailler en Suisse, où leur salaire est parfois multiplié par trois.

Des négociations concrètes et à visée opérationnelle sont en cours. La conclusion de cet accord constituera un progrès pour le territoire, mais il conviendra auparavant de faire converger des intérêts réciproques.

Après la finalisation des conventions sur l'aide médicale d'urgence, les travaux se concentrent désormais sur la mise en place d'un observatoire transfrontalier réunissant le Luxembourg, la Suisse et la Belgique autour de la question de la simplification des modalités de prise en charge et des projets de contrats locaux de santé transfrontaliers. L'ARS travaille en lien étroit avec les autorités préfectorales, les collectivités locales, l'assurance maladie, Santé publique France et les établissements de santé sur ces différents sujets. Dans le cadre du schéma régional de santé 2023-2028, qui est en cours de finalisation, nous tracerons de nouvelles perspectives concernant ce volet transfrontalier : il faudra faudra notamment faire une analyse de la démographie des professionnels de santé de part et d'autre de la frontière, afin d'envisager un plan d'actions précis du territoire, particulièrement avec l'Allemagne, État avec lequel la collaboration se déroule favorablement dans le cadre de l'Union européenne.

Comme l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements sanitaires, des services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement sanitaire ou à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les personnels en catégorie active relevant des corps placés en voie d'extinction bénéficient du complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros net par mois.

Les agents relevant des corps de la catégorie active sont très majoritairement en fin de carrière et se trouvent sur les échelons les plus élevés de leur grille indiciaire. Par contraste, les personnels relevant des corps de la catégorie sédentaire sont majoritairement en début de carrière : ils sont donc peu nombreux à bénéficier des échelons élevés de leur grille indiciaire.

le non-remplacement d'un des deux médecins nécessaires au bon fonctionnement du service des urgences. Certes, un seul médecin ne peut pas à la fois prendre en charge les urgences vitales dans les services, les hospitalisations non programmées et assurer les opérations du Smur. Cette prise en charge, lorsque l'un des médecins est en intervention dans le cadre du Smur, est en effet possible temporairement, mais elle ne peut devenir la règle- nous en convenons. Pour autant, la seule fermeture du Smur est-elle une réponse acceptable à l'absence de l'un des deux médecins ? Ne pose-t-elle pas à terme la question de la pérennité du service des urgences indispensable aux habitants de ce territoire ? D'autant plus que ce dysfonctionnement n'est pas le seul que l'on recense : depuis plusieurs années déjà, l'hôpital d'Orthez ne cesse de dénoncer le manque de personnel, notamment l'absence d'un poste d'infirmier d'accueil, qui empêche une prise en charge adaptée des patients.

La doctrine nationale prévoit, en présence d'un seul médecin urgentiste, et ce afin de garantir la continuité de l'accès aux soins, la mise en place d'un mode de fonctionnement gradué privilégiant le maintien du Smur, et la mise en oeuvre d'un accès régulé aux urgences, le centre 15. L'ARS de Nouvelle-Aquitaine, dans le respect de cette doctrine, s'attache à coconstruire une organisation territoriale des urgences visant à répondre à la problématique des ressources médicales, et à définir un mode de fonctionnement commun solidaire en cas d'absence inopinée de praticiens.

et de la prévention. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur la nécessité de soutenir les élus locaux dans les communes rurales confrontées à des problématiques de démographie médicale. d'illustration, le département de la Mayenne, dont je suis élu, ne compte plus aujourd'hui que 6,2 généralistes pour 10 000 habitants. Certains services d'urgence et de maternité sont contraints de fermer par intermittence. Beaucoup trop de patients ne parviennent pas à trouver de médecin traitant. Les médecins spécialistes, dentistes et gynécologues particulièrement, se font rares, sans parler des médecins du travail dont le rôle est pourtant si essentiel pour nos travailleurs. Les infirmières libérales voient quant à elles leurs conditions de travail se dégrader. Dans ce contexte, la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, dite Rist, a permis quelques avancées. Ce n'est toutefois pas suffisant.

Alors que la population vieillit et que les pathologies chroniques sont de plus en plus récurrentes, ces maisons sont essentielles pour assurer la bonne coordination des soins et la prise en charge pluridisciplinaire du patient. Elles essaiment partout sur le territoire, mais, malgré leur fort engagement en la matière, nos élus

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, notre priorité est de lutter contre toutes les inégalités de santé, et de proposer pour tous, et partout en France, un accès à des soins adaptés et de qualité. Créer les conditions d'une attractivité rénovée de nos territoires, pour que les professionnels viennent s'y installer, et surtout, y restent pour mener des projets personnels et professionnels de long terme, nécessite une mobilisation de l'État, comme de tous les acteurs locaux, au premier rang desquels les élus des territoires ruraux, dont nous ne sous-estimons pas l'engagement quotidien et auxquels le Gouvernement s'attache à donner les outils nécessaires. Les efforts que nous menons avec les ARS dans tous les territoires

des soins médicaux et de rééducation (SMR), en particulier dans le contexte de l'Île-de-France. La réforme du financement, qui était souhaitée et qui a été longuement concertée, n'est pas encore au point

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, comme vous le soulignez, les premières études d'impact concernant cette réforme ont pu faire apparaître des pertes de ressources pour certains établissements SMR de la région Île-de-France. Toutefois, il convient de souligner qu'il s'agit de projections qui ne sont en rien figées. Elles ont justement pour finalité de servir de base de travail et doivent permettre l'ajustement des paramètres associés dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles modalités de financement. Une nouvelle version amendée est ainsi en préparation, laquelle devrait permettre de corriger les distorsions les plus manifestes tout en donnant davantage de visibilité pluriannuelle aux acteurs. Par ailleurs, si l'application de la réforme est bien prévue pour le 1 juillet 2023, il est important de rappeler que le nouveau modèle n'est pas d'application immédiate. Ainsi, afin de simplifier et de stabiliser la campagne budgétaire pour l'ensemble des acteurs, les vecteurs actuels de financement seront maintenus jusqu'à la fin de l'année, notamment les prix de journée pour le ex-OQN (ex-objectif quantifié national). L'application des impacts de la réforme sera faite, selon une méthodologie partagée avec les fédérations d'établissements SMR et les agences régionales de santé la reprise des crédits déjà alloués aux établissements durant la campagne au titre de l'exercice 2023. Un mécanisme de transition visant par ailleurs à amortir les impacts de la réforme et à sécuriser les trajectoires financières des établissements est prévu sur trois ans. Cette période doit justement permettre d'affiner les nouvelles modalités de financement afin de prendre en compte dans leur complexité l'ensemble des enjeux de filières et de territoires pour les SMR. Concernant les surcoûts induits par les conditions propres à l'Île-de-France, le coefficient géographique sera bien pris en compte dès l'application de la réforme. Concernant les activités spécifiques dont vous soulignez, à juste titre, la valeur ajoutée dans la prise en charge des patients, mais également les surcoûts spécifiques au regard de la charge en soins associée, des groupes de travail nationaux sont prévus afin de s'assurer de leur juste prise en compte dans le modèle. Des travaux sont encore en cours sur les grilles tarifaires des séjours, qui seront applicables dans le futur modèle. Ils ont vocation à identifier les situations qui apparaissent de manière systématique insuffisamment valorisées et qui doivent faire l'objet d'ajustements en amont de la publication des prochains tarifs.

Heureusement qu'une période de glissement avant l'application de la nouvelle réforme aura lieu. Je ne peux que former le voeu que la discussion se conclue positivement pour tout le monde.

alors même que le taux d'élèves en situation de handicap psychique est de dix points supérieur à la moyenne de l'académie. Ce décalage entre les besoins de la population et la réponse publique laisse place à des situations dramatiques pour les jeunes concernés. Votre objectif d'une école inclusive est louable, mais se heurte à la réalité de l'accompagnement en France. Malheureusement, vous avez fait le choix de fermer un nombre important de places dans les différentes structures spécialisées avant même de vous assurer que la prise en charge de ces élèves était réalisable dans de bonnes conditions dans le système classique. Ainsi, de nombreuses familles ne disposent d'aucune bonne solution : l'accueil dans des structures classiques est souvent très inadapté. Face à cela, une centaine de jeunes Charentais sans solution sont déscolarisés. Ces jeunes sont pour la plupart sur des listes d'attente longues de deux ans pour un accès en Itep et de (IME). Pour les jeunes atteints de troubles autistiques, l'attente peut aller jusqu'à six ans. Par ailleurs, cet embouteillage est aggravé par le manque de places d'accueil pour les personnes majeures en handicap qui sont accueillies dans les IME. Les enfants de la République ont tous le droit à l'école. L'idéal républicain n'en est plus un si des élèves sont exclus du système scolaire sur le fondement de leur handicap. Madame la ministre, quelle réponse entendez-vous apporter à ces familles maltraitées et à ces enfants ? Comment comptez-vous créer de nouvelles places dans les établissements médico-sociaux Itep et IME en Charente ?

Ces chiffres recouvrent des réalités très diverses. Il est vrai que certaines familles doivent attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant de trouver une situation adaptée. Ce n'est pas acceptable. Pour autant,

L'offre de répit ainsi qu'un accompagnement spécifique pour les enfants en situation de handicap relevant de l'aide sociale à l'enfance sont également développés. Cela a été possible grâce à l'engagement du conseil départemental aux côtés de l'ARS. Nous voulons aller plus loin, notamment pour les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton, pour les territoires en zone blanche et pour les enfants et adultes autistes. Lors de la Conférence nationale du handicap du 26 avril dernier, le Président de la République a présenté soixante-dix mesures dont la création de 50 000 nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, adaptées au parcours de chacun et dans le respect de ses choix. Concernant la question des plus jeunes et de leur scolarisation, mon collègue Pap Ndiaye et moi-même travaillons à ce que l'école s'adapte à tous les élèves en situation de handicap et non l'inverse. Dans les mois à venir, la transformation des établissements pour enfants en dispositifs et plateformes ouverts, plus fluides, permettra de répondre aux différentes situations évoquées. Madame la sénatrice, notre ambition est l'exercice de tous les droits pour tous les citoyens.

Ce dernier élargit l'accès à cette prestation aux personnes atteintes d'un handicap psychique, cognitif, mental ou de troubles du neuro-développement et inclut la prise en compte des besoins spécifiques des personnes souffrant de déficience auditive et visuelle. ce texte constitue une avancée en matière de reconnaissance et de compensation pour les personnes en situation de handicap atteintes de ces pathologies, et c'est pourquoi le département de la Haute-Loire s'inscrit pleinement dans cette prise en compte. département, selon les premières estimations, cette nouvelle extension de la PCH entraînera un surcoût annuel compris entre 700 000 et 2,5 millions d'euros, compte tenu du nombre de dossiers de nouveaux bénéficiaires. Pour l'année 2022, la compensation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) était portée à 3,9 millions d'euros pour un budget de la PCH à domicile et en établissement s'élevant à 7,7 millions d'euros. Les dépenses liées à la mise en oeuvre de la PCH et à ses ajustements successifs sont venues grever chaque année les dépenses à un rythme et à une échelle que les concours attribués par la CNSA ne couvrent plus. Par conséquent, au vu de l'accroissement du nombre de dossiers, je souhaiterais savoir, madame la ministre, si le concours de la CNSA versé au département au titre de la PCH sera notablement revu afin de compenser ces prévisions de dépenses et ce dans l'optique de trouver un juste équilibre entre les enjeux de compensation du handicap auxquels notre territoire souscrit pleinement et la préservation budgétaire des collectivités territoriales. La parole Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur, comme pour la réponse précédente, Mme Darrieussecq m'a demandé de vous fournir les éléments suivants, en réponse à votre interrogation. Vous avez bien voulu nous interroger sur la révision du concours de la CNSA au titre de la PCH versée aux départements. La CNSA finance par concours plusieurs dépenses des conseils départementaux en lien avec leur mission dans le cadre de leurs compétences sociales

handicapées (MDPH), et d'autres dépenses encore. S'agissant de la PCH, les concours de la CNSA ont augmenté, passant de 510 millions d'euros en 2009 à 637 millions d'euros en 2021, soit une augmentation d'un quart. Concernant la PCH pour les personnes avec des troubles psychiques, intellectuels, cognitifs ou des troubles du neuro-développement, cela est effectif depuis le 1 janvier dernier. Le dispositif est donc en train de se déployer et de monter en puissance. Notre responsabilité conjointe entre État et départements est désormais de s'assurer que cette avancée majeure bénéficie concrètement aux personnes qui sont concernées sur le terrain. Je vous y sais attentif et vous en remercie. Lors des travaux préparatoires, nous nous sommes engagés à suivre de près l'évolution de ces dépenses induites par cette PCH « psy » ainsi que celle des modalités et des montants de la couverture par la branche autonomie. Enfin, depuis l'année dernière, la mise en place d'un comité des financeurs avec Départements de France a créé une instance de dialogue régulière entre le Gouvernement et les conseils départementaux sur les sujets de compensation des politiques d'autonomie. Cela assure un suivi partagé et objectivé des évolutions de dépenses. Monsieur le sénateur, soyez assuré que le Gouvernement est particulièrement attentif aux enjeux de ces dépenses de solidarité et de compensation du handicap dans les territoires.

ils sont très loin de couvrir les 2,5 euros de coût de production et de rémunérer les producteurs. Le retrait de la production en stock, s'il se met en place avec les programmes opérationnels, ne concernera que les agriculteurs en organisation de producteurs ou en coopérative. Les autres seront exclus. Il y a urgence à additionner ce dispositif de retrait avec des mesures de fond d'allègement de charges. Ce type de demande est régulièrement mis en place pour les productions en crise. Le verger de noix est tout de même le deuxième verger de France. Une fois ces mesures prises, il faut faire appliquer la préférence communautaire et imposer les clauses miroirs pour l'importation de produits qui ne respectent pas nos normes sociales, sanitaires et environnementales. De plus, une campagne de communication sur les bienfaits diététiques de la noix doit s'opérer. Si la consommation passait de 200 à 400 grammes par an et par Français, la crise serait en partie résolue.

exemplaires et doivent être défendus. Les recommandations de la Cour des comptes sont irresponsables dans la situation que vit notre agriculture. Cela est vécu comme une véritable blessure par nos éleveurs. Ne réservons pas à l'agriculture le traitement infligé à l'industrie

Ce dispositif a été activé par FranceAgriMer et les organisations professionnelles peuvent se saisir de cet outil de gestion de crise pour faire du retrait et réguler le marché domestique. Deuxièmement, il faut mettre en valeur le produit. Cela doit se faire par une communication à l'intérieur de nos frontières, y compris avec la restauration collective ou la grande distribution, pour faire en sorte de déstocker. Cela passe aussi par un travail sur l'export, comme vous l'avez mentionné. Troisièmement, il faut aussi faire évoluer la production et lui offrir de nouveaux marchés : c'est toute l'ambition du plan de souveraineté Fruits et Légumes que nous avons lancé pour répondre aux enjeux de compétitivité et de planification écologique.

2023. Sur la question de l'élevage et du rapport de la Cour des comptes, Marc Fesneau a, devant le Sénat, réaffirmé avec force son soutien à nos éleveurs. La Première ministre a également eu l'occasion de le faire au nom du Gouvernement devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Oui, nous sommes fiers de nos éleveurs ; oui, nous avons besoin d'élevage pour notre souveraineté alimentaire, mais aussi pour toutes ses externalités positives. C'est non pas contre, mais bien avec nos éleveurs que nous mènerons les transitions. La parole est à M. Cédric Perrin, et de la fonction publiques. La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot affecte 5 000 à 7 000 patients en France. Aujourd'hui même, trois nouveaux cas ont été déclarés, ce qui fait que la maladie est de moins en moins rare. et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a représenté un véritable tournant, l'égalité n'est pas encore au rendez-vous, comme en témoigne l'exemple qui suit. Les différents dispositifs de congé spécial de la fonction publique territoriale, en particulier ceux dont peut bénéficier la personne fonctionnaire atteinte de la maladie de Charcot, peuvent en effet susciter des En vertu de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire peut être placé en congé de longue durée s'il est atteint par l'une des maladies suivantes : cancer, déficit immunitaire, maladie mentale, tuberculose et poliomyélite. Cela exclut la personne touchée par la maladie de Charcot. Le congé de longue durée permet au fonctionnaire de conserver pendant trois ans l'intégralité de son salaire et la moitié de celui-ci les deux années suivantes. En revanche, la personne fonctionnaire atteinte par la maladie de Charcot ne peut prétendre qu'au congé de longue maladie. Elle perçoit alors l'intégralité de son traitement pendant un an seulement et la moitié les deux années suivantes. Ce congé est moins avantageux d'u point de vue financier alors même que les perspectives d'évolution de cette maladie sont similaires à celles des pathologies listées précédemment. Cette maladie dégénérative ne permettra nullement une reprise, même ponctuelle, de l'activité professionnelle. Madame la ministre, quelles sont selon vous les raisons qui pourraient justifier une telle différence de traitement ? J'imagine facilement que vous n'en trouverez aucune, d'où ma seconde question

ne peut bénéficier du congé de longue durée prévu aux articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique. Il peut néanmoins prétendre à l'octroi d'un congé de longue maladie de trois ans maximum, dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement, en cas d'affection grave nécessitant un traitement et des soins prolongés. Contrairement au congé de longue durée, qui ne peut être octroyé qu'une seule fois par affection, le congé de longue maladie est par ailleurs renouvelable si le fonctionnaire a repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. En outre, si, pendant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, le fonctionnaire territorial n'a pas bénéficié de plus d'un an de congé de longue maladie, il continue à percevoir un plein traitement. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est rouvert intégralement quatre ans après l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Dans le cadre du plan d'accompagnement des maladies chroniques qu'il a lancé le 1 juin dernier, le ministre Stanislas Guerini a fait de l'amélioration de la protection des agents publics malades sa priorité. Des évolutions relatives aux arrêts maladie longs seront présentées dans le cadre des négociations sur la prévoyance dans la fonction publique, qui doivent qui doivent aboutir d'ici à mi-juillet.

Si, en apparence, l'idée peut paraître adaptée aux besoins d'accompagnement des élus locaux, notamment ruraux, les conditions d'application le sont beaucoup moins.

liés, par exemple, aux situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils peuvent se trouver. Si je résume, le premier venu peut donc candidater pour donner des conseils juridiques à des élus locaux contre une indemnité quant à elle plafonnée à 80 euros, quels que soient la mission effectuée et le temps de travail s'y rapportant. rédacteurs de ce décret manquent de bon sens. Dans les territoires ruraux, dans lesquels les profils attendus peuvent manquer et où les consultations risquent d'être peu nombreuses, les conditions actuelles de désignation d'un référent déontologue semblent irréalistes, voire inopérantes. Que compte donc faire le Gouvernement pour clarifier et simplifier ce dispositif-

d'un amendement parlementaire lors de la discussion de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a fait l'objet d'une large concertation avec les associations d'élus. Le décret en Conseil d'État du 6 décembre 2022 en est la traduction avec la double préoccupation, d'une part, de garantir l'impartialité de ce référent qui doit conseiller utilement l'élu local sur le respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local, d'autre part, de laisser une grande souplesse aux collectivités territoriales pour la mise en place du référent. En outre, le décret précité n'est entré en vigueur que le 1 juin 2023, soit près d'un an et demi après la loi du 21 février 2022. Le Gouvernement n'a pas prévu de revenir sur cette mesure importante pour accompagner les élus dans leur mandat. Il s'agit toutefois d'un dispositif souple : le décret tend à ce que l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales ou syndicat mixte désigne le référent déontologue tout en permettant la désignation d'un même référent par plusieurs collectivités, groupements de collectivités ou syndicats mixtes, par délibérations concordantes. Un guide, qui fait l'objet d'échanges avec les associations d'élus, sera prochainement diffusé par la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité pour appuyer les collectivités dans la mise en oeuvre de ce dispositif. La parole

avons à organiser la mise en place de ce déontologue. Il n'y a pas de solution : les 80 euros de rémunération ne sont pas attractifs pour l'éventuel impétrant. Je pense donc qu'il faudrait un délégué par département. J'attends avec beaucoup d'impatience la circulaire dont vous venez de me parler.

En 2019, une mission d'information sénatoriale à laquelle j'ai participé a alerté sur l'urgence qu'il y avait à décréter un véritable plan Marshall pour les ponts. En juin 2022,

Conscients de l'urgence et de l'enjeu, les sénateurs ne cessent d'essayer, lors des projets de loi de finances, de prévoir des crédits affectés aux travaux dans des proportions qui ne soient pas ridicules ... En général, ces tentatives sont peu suivies Concrètement, à l'heure actuelle, il y a en France, presque dans chaque commune, y compris les plus petites, des ponts qui ont besoin urgemment de travaux, parfois lourds. Face à cette urgence, les maires bénéficient dans le meilleur des cas de la Ils n'ont pas la possibilité de trouver des cofinancements et sont rarement en situation de financer les 70 % restant à leur charge. Madame la secrétaire d'État, face à cette situation, que compte faire le Gouvernement ? La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Pour répondre à ce besoin d'accompagnement, le Gouvernement a proposé aux petites communes de bénéficier gratuitement d'un recensement de leurs ouvrages et d'un premier diagnostic de ceux présentant des désordres : il s'agit du programme national Ponts.

Plus de 11 000 communes ont demandé à en bénéficier. Le programme est désormais proche de son terme et plus de 45 000 ouvrages ont été ainsi recensés. Fort de ce succès, le Gouvernement a décidé en avril dernier l'extension du programme à 4 000 nouvelles communes en mobilisant une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros. Cette enveloppe permettra également d'offrir une nouvelle occasion aux communes éligibles au premier programme qui n'ont pas candidaté et qui souhaiteraient finalement le faire. Par ailleurs, une aide au financement des travaux sera également proposée aux communes éligibles au programme national Ponts. Le dispositif sera présenté à l'été 2023. Vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement a été particulièrement attentif aux alertes du Sénat et se tient résolument aux côtés des collectivités.

à notre connaissance, ou en tout cas ne sont pas clairs : nous n'avons pas de réponses. Je voudrais être certaine que le Cerema aura vraiment une feuille de route qui permettra de travailler efficacement. Pour élargir un peu le débat, outre les moyens financiers, de quels moyens humains disposerons-nous ? En effet, je signale au passage que la France forme à l'heure actuelle 30 000 ingénieurs alors qu'il en faudrait 40 000 et que le pic de dégradation des ouvrages d'art est devant nous. Il faut impérativement des choix stratégiques forts face à ce qui est, en fait, une catastrophe annoncée. La parole est à Mme Patricia Demas,

pour atteindre l'objectif très ambitieux de la neutralité carbone en 2050. Si l'on ne peut que louer l'intention nourrie au travers de ce dispositif national, on comprend néanmoins difficilement que la forêt méditerranéenne en soit écartée. La région Sud est la deuxième région de France en matière de surface boisée ; plus de 60 % du territoire des Alpes-Maritimes sont recouverts de forêt. Or ses spécificités ne sont pas reconnues. La croissance plus lente de ses arbres n'est malheureusement pas prise en compte dans le dispositif national et les pénalités infligées en matière de risque incendie l'excluent de projets d'entretien ou de reconstitution. (Giec) indique par ailleurs un accroissement des températures et des périodes de sécheresse plus fort pour la région méditerranéenne que dans le reste du territoire national, provoquant un dépérissement des peuplements forestiers qui a des conséquences sur la quasi-totalité des espèces. Les enjeux sont forts. Madame la secrétaire d'État, il faudrait assouplir les critères d'éligibilité pour que la forêt méditerranéenne soit pleinement admissible au label Bas-carbone, d'autant que, localement, la demande des acteurs économiques y est forte. Les Alpes-Maritimes sont prêtes à innover dans la méthode et à devenir un territoire pilote, entre autres avec la sylviculture du pin d'Alep. Dans ce contexte, je me permets d'insister sur la nécessité d'autoriser l'inclusion de la forêt méditerranéenne dans le dispositif label Bas-carbone

Le fonds vert, annoncé en août 2022 par la Première ministre, a pour ambition d'accompagner les collectivités dans leurs projets en lien avec la transition écologique des territoires. Il est doté de 2 milliards d'euros et répond à un triple objectif : renforcer la performance environnementale, adapter les territoires au changement climatique et améliorer le cadre de vie. Le déploiement du fonds vert repose sur une répartition des crédits entre régions afin de répondre aux enjeux spécifiques des territoires. La Guyane a en effet reçu une enveloppe de 9 millions d'euros qui permettra de mettre en oeuvre divers projets au service de la transition écologique. Comme dans la plupart des autres régions, l'aide demandée au titre du fonds vert excède l'enveloppe déléguée. Ce constat reflète la forte demande des collectivités et leur volonté de participer à l'effort collectif qu'exige la transition écologique : 12 200 dossiers ont été déposés, et 4,1 milliards d'euros ont été demandés pour un total de 17,5 milliards d'euros d'investissement local. Le fonds vert joue donc bien son rôle d'accélérateur de la transition écologique dans les territoires, et je salue votre intérêt pour le dispositif. Si la demande globale de financement, au niveau national, se situe à hauteur de 24 % du montant total des projets,

L'exercice 2023 a constitué la première année du déploiement du fonds vert, et l'intégralité des crédits devrait être engagée d'ici à la fin de l'année pour soutenir un grand nombre de projets, en métropole et dans les territoires

Ces derniers sont tout à fait prêts à s'engager dans une démarche plus vertueuse, mais des freins restent à lever. En effet, à ce jour, le secteur des travaux publics se heurte en particulier à trois freins principaux : l'offre, le temps et le coût. L'offre de véhicules est en cours de structuration, tandis que les différentes infrastructures de recharge sont naissantes et ne permettent pas, à ce jour, à ces entreprises de répondre au calendrier de la ZFE. Il convient également de prendre en compte l'aspect financier, car ces entreprises sont touchées de plein fouet par l'inflation, et ce après trois années post-covid difficiles. Cette nouvelle obligation imposée par la loi fait peser sur cette profession des contraintes budgétaires élevées. Je vous l'assure, madame la secrétaire d'État, toute la filière est pleinement mobilisée autour des enjeux de la mobilité, mais il est aujourd'hui nécessaire d'adapter les contraintes et le calendrier aux réalités économiques de ces entreprises et à leur capacité je souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour aider ces entreprises des travaux publics, soucieuses de s'inscrire dans cette démarche écologique visant à protéger les populations de la pollution.

mobilité sont un outil aux mains des collectivités pour améliorer la qualité de l'air. La mise en place des ZFE répond à une nécessité de santé publique, car plus de 40 000 décès sont imputables chaque année à la pollution atmosphérique d'après Santé publique France. Le coût annuel pour la société française de la pollution de l'air est estimé à 100 Je tiens à préciser que, parmi les territoires devant mettre en place une ZFE, seules les agglomérations qui dépassent de façon régulière les valeurs limites en matière de qualité de l'air sont tenues de respecter un calendrier de restrictions à la circulation de certains véhicules, en fonction de leur vignette Crit'Air. Ces restrictions concernent les voitures de particuliers, et ne s'appliquent pas aux poids lourds ou aux véhicules utilitaires légers. Les autres agglomérations décident, en fonction du contexte local, de la temporalité des restrictions imposées, des catégories de véhicules visées et des éventuelles dérogations. Christophe Béchu a souhaité renforcer les échanges avec les collectivités pour réunir des conditions favorables au déploiement des ZFE, notamment par le biais de la mise en place d'un comité ministériel de suivi des ZFE en octobre 2022 et la mise en oeuvre d'un comité de concertation sur les ZFE. Ce dernier, piloté depuis janvier 2023 par Jean-Luc Moudenc et Anne-Marie Jean, doit établir des propositions très opérationnelles pour harmoniser les caractéristiques des ZFE, assurer leur acceptabilité sociale et accompagner les usagers. Le dispositif des ZFE doit par ailleurs s'accompagner d'un verdissement du parc, et des aides de l'État existent pour accompagner les professionnels dans cette transition.

Madame la secrétaire d'État, il me semble nécessaire de recueillir aujourd'hui votre position sur la problématique des reprises de friches industrielles dans les territoires, notamment dans les communes rurales, confrontées aux objectifs croisés du zéro artificialisation nette (ZAN), de revitalisation urbaine et de territorialisation et de la nécessaire approche pragmatique avec laquelle ce sujet doit être abordé.

La mise en place d'un fonds par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, pour financer des opérations de recyclage des friches et la transformation de foncier déjà artificialisé, témoigne d'ailleurs de l'importance accordée au sujet par le Gouvernement. Or la complexité du réinvestissement des friches contraint régulièrement les territoires à abandonner certains projets de réhabilitation pourtant validés par un architecte urbaniste et le conseil municipal, comme c'est le cas dans la Sarthe, les moyens d'organisation de ce desserte, flux de circulation généré -nécessitant un ajustement de son périmètre. Il serait donc judicieux d'acter, au-delà des caractéristiques de la friche en elle-même, la prise en compte des spécificités des territoires et de la nature même du projet pour poser les enjeux de développement du territoire et ainsi définir la vocation du site dans cette trajectoire. À cette fin, je souhaiterais connaître votre position concernant une éventuelle approche en souplesse des caractéristiques propres à la friche, et particulièrement de son périmètre, ainsi que les mesures pouvant être mises en place, notamment au niveau des documents de planification,

de revitalisation urbaine et de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le préfet Rollon Mouchel-Blaisot a été chargé par le Gouvernement d'une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel. la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience. Les modalités d'application de cette définition seront définies par décret. Conscients de la complexité opérationnelle d'un projet de reconversion d'une friche, l'État et ses opérateurs ont développé des outils pour accompagner les porteurs de projets et les collectivités territoriales, tels que l'outil, qui vise à mieux connaître le site de friche urbaine identifié, les acteurs et les outils pour lancer les premières études et aider dans la recherche de financements.

La loi Climat et résilience a introduit un bonus de constructibilité de 30 %, pour faciliter l'équilibre économique de l'opération, avec une plus grande densité des projets réalisés dans les friches. Enfin, l'État alloue des subventions en faveur du recyclage des friches : 750 millions d'euros pour la période 2021-2022 dans le cadre du fonds Friches, au bénéfice de 1 382 projets lauréats. Ce fonds a été pérennisé en 2023 grâce au fonds vert, doté de 2 milliards d'euros, qui suscite un fort intérêt, avec plus d'un millier de projets de recyclage des friches en cours d'instruction. La parole est à M. Frédéric Marchand, Madame la secrétaire d'État, avec 4 345 habitants recensés en 2018, Avesnes-sur-Helpe est la sous-préfecture la moins peuplée du Nord. L'évolution démographique depuis 1968 montre une baisse constante atteignant une perte d'habitants de 30 %. La commune connaît une réelle problématique de baisse de sa population, en partie liée à sa problématique de logement. En effet, depuis 2014, elle est sortie du dispositif de la politique de la ville et des contrats urbains de cohésion sociale Un programme d'action à destination des publics spécifiques dans les quartiers prioritaires permettait de niveler les différences sociales sur des champs thématiques divers, tels que l'éducation, la culture, la prévention de la délinquance, la santé, et bien d'autres domaines. Cependant, aucun programme de rénovation de l'habitat du type opération programmée d'amélioration de l'habitat (Opah) n'a été activé par la municipalité en charge du dossier à l'époque, ce qui est aujourd'hui fort préjudiciable à la qualité et à la diversité des logements sur cette commune. Il est d'ailleurs à relever une très forte prédominance du parc privé, issu majoritairement de maisons individuelles divisées en appartements, ce qui explique une vacance préoccupante. Par ailleurs, la commune doit également faire face à un taux très élevé de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL) supérieur de 16 points au ratio départemental. Le parc social, majoritairement antérieur à 1970, est vieillissant. Il est de surcroît mal adapté aux typologies familiales actuelles, avec la prédominance de familles monoparentales et de familles moins nombreuses. Depuis 2020, le nouveau maire et son équipe ont engagé des politiques volontaristes, en s'appuyant notamment sur le pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache. Les résultats de ce dynamisme sont au rendez-vous, puisque la ville d'Avesnes-sur-Helpe est lauréate du programme Petites villes de demain et signataire, en novembre 2022, d'une opération de requalification territoriale. Le projet de la commune repose sur la mise en valeur et la restauration du patrimoine architectural, le développement du tourisme, le soutien au commerce local de proximité et l'instauration d'un programme d'intervention sur l'habitat, pour placer la ville au centre de la dynamique territoriale. Autour d'axes forts, la ville oeuvre à un projet global environnemental, patrimonial, éducatif, culturel et social. Cet outil puissant doit être un levier, avec le concours d'une opération de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, pour redimensionner les quartiers de la commune en situation de fragilité sociale.

loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. L'article 5 de cette loi prévoit que les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par un nombre par un nombre minimal d'habitants et un écart de développement économique et social apprécié par le critère de revenu par habitant. Le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 a précisé la méthodologie de définition des quartiers pour la France métropolitaine. Conformément au 1° de l'article 2-1 du décret, « les territoires urbains sont les unités urbaines définies par l'Insee ayant une population d'au moins 10 000 habitants ». Selon la base des unités urbaines 2020 de l'Insee, la commune d'Avesnes-sur-Helpe appartient à une unité urbaine de moins de 10 000 habitants. Des concertations locales se tiennent actuellement sous l'égide des préfets pour déterminer les contours des nouveaux quartiers prioritaires, en respectant les critères actualisés de pauvreté et de population. Le Gouvernement souhaite toutefois redonner la capacité aux acteurs locaux d'intervenir dans certains quartiers qui ne répondraient pas aux conditions fixées par la loi, par exemple des poches de pauvreté ou des quartiers qui décrochent brutalement, pour adapter la réponse publique à la réalité locale. en cours de la politique de la ville sera ainsi l'occasion de donner une nouvelle ambition à cette politique, nourrie de la participation des habitants des quartiers et des dynamiques positives enclenchées. Je sais que vous devez, demain, rencontrer M. le ministre avec la maire d'Avesnes-sur-Helpe. Il sera

qui s'affranchirait des enjeux essentiels à l'équilibre et à la vie de nos territoires, que sont la rénovation et la revitalisation de nos villages et de nos bourgs. Les élus sont tous conscients qu'il est essentiel de concilier l'atteinte des objectifs de sobriété foncière avec celui du développement des territoires ruraux, afin de répondre aux défis environnementaux et sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est être de simples exécutants de l'application rigoureuse des textes. Ils veulent être en mesure de coconstruire leur développement, d'oeuvrer à l'aménagement de leur territoire et d'être en mesure d'opérer des choix stratégiques, en concertation

bâti vacant dans les communes rurales, intégrant des moyens financiers, un accompagnement en ingénierie, des outils juridiques facilitant le changement de destination du bâti, notamment agricole, l'inscription dans la loi d'un « droit au projet » autorisant le portage de projets d'intérêt communal ou multicommunal. de permettre plus à ceux qui ont artificialisé moins, c'est-à-dire d'assurer une garantie rurale. Il convient enfin d'intégrer une juste prise en compte des projets d'envergure nationale n'impactant pas les territoires qui n'en auront aucune retombée. Aussi, j'espère que le Gouvernement tiendra sa promesse de poursuivre la discussion sur la base du texte adopté par le Sénat et qu'il sera à l'écoute de tous nos élus locaux, acteurs des territoires, lors de l'examen à l'Assemblée nationale les 21 et 22 juin prochain de la proposition de loi

chaque année, 21 000 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers sont consommés en moyenne en France. Les conséquences sont écologiques, avec un impact direct sur l'érosion de la biodiversité et le stockage de carbone, mais aussi socioéconomiques. La France s'est donc fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour la période 2021-2031.

grands projets d'intérêt national. La proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, déposée par les sénateurs Valérie Létard et Jean-Baptiste Blanc, a été adoptée le 16 mars 2023 par la Haute Assemblée. Nous tenons ici à saluer l'engagement du Sénat pour faire évoluer les dispositions relatives au ZAN, afin de permettre davantage de souplesse dans sa mise en oeuvre au niveau des territoires. La proposition de loi sénatoriale demeure, pour le Gouvernement, le véhicule privilégié pour faire évoluer le dispositif du ZAN.

L'objectif du Gouvernement est de parvenir, par la concertation avec les associations d'élus locaux et le dialogue avec les deux chambres du Parlement, à l'adoption d'un texte consensuel, conforme aux grandes orientations résumées dans le discours de la Première ministre. Les questions que vous soulevez sont au coeur des débats qui animeront le Parlement ces prochaines semaines. La parole

face à l'urgence écologique et à l'impératif de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, le ferroviaire est la solution incontournable. Les deux lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (Polt) et Paris-Clermont-Ferrand desservent près du quart du territoire national, cinq régions et dix millions d'habitants. Ce sont des axes reconnus comme structurants par l'État. L'objectif est bien d'augmenter le nombre de voyageurs, même de le doubler, selon la SNCF, et de garantir un service plus équitable plus équitable aux usagers des territoires desservis. Pour rappel, un Paris-Marseille dure trois heures, un Paris-Bordeaux, deux heures, alors qu'un Paris-Cahors dure jusqu'à six heures, ce qui situe Cahors, en quelque sorte, bien au-delà de la frontière espagnole.

important, permettant notamment d'accroître l'ambition du schéma directeur, soit quatorze allers-retours au lieu de onze et un gain de temps de 35 minutes sur le Paris-Toulouse. Pour autant, nous tenons absolument au programme minimum du schéma directeur pour 2025, à réaliser sans faute. La Première ministre a déclaré non seulement que « moderniser se traduira par davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs », mais aussi que « notre stratégie doit bénéficier à tous les Français, où qu'ils vivent, des petites communes jusqu'aux grandes métropoles ». Autrement dit, nous correspondons exactement au coeur de cible du plan d'avenir. Nous avons en effet besoin d'un avenir ferroviaire, en tant que véritables oubliés du rail. Les habitants des territoires desservis par la ligne Polt doivent être une des priorités du plan annoncé par la Première ministre. Cette ligne doit être soutenue de manière significative dès 2023. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, je vous demande de préciser quelle sera, sur les 100 milliards

! La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice Préville, je vous confirme l'attention particulière que le Gouvernement porte à la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, qui constitue un axe nord-sud stratégique pour notre pays. Cette ligne bénéficiera d'investissements significatifs de la part de l'État : arrivée d'un nouveau matériel roulant, dont le financement s'élève à 450 millions d'euros, et programme de modernisation visant à améliorer les performances de la ligne d'ici à 2026, avec un investissement de l'État à hauteur de 257 millions d'euros. Par ailleurs, des travaux de régénération entièrement financés par SNCF Réseau sont réalisés jusqu'en 2025, afin de remettre à niveau l'infrastructure, pour un montant total de 1,6 milliard d'euros. Ces travaux avancent conformément à la trajectoire prévue. Lors de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, la Première ministre a indiqué s'appuyer sur le scénario « planification écologique », dans le cadre des arbitrages à venir relatifs au plan d'investissement dans les infrastructures de transports. Naturellement, l'ensemble de ces investissements, actés dans le schéma directeur de la ligne Polt, sont intégrés dans la trajectoire ambitieuse d'investissements annoncée par la Première ministre. Afin d'assurer un suivi plus régulier associant les parties prenantes, le ministre délégué chargé des transports a demandé à la SNCF la mise en place d'un groupe de travail technique se réunissant à fréquence trimestrielle et se concentrant sur les améliorations de la qualité de service. Je vous confirme ainsi l'engagement du Gouvernement pour l'amélioration de la robustesse et de la qualité de service

Madame la secrétaire d'État, des collectifs, des associations, des élus, des riverains se mobilisent pour alerter sur un problème de santé publique. Il s'agit de la pollution sonore aux abords de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont les nuisances se répercutent sur le quotidien des habitantes et habitants des alentours. Le bruit est la seconde menace pour la santé environnementale, après la pollution atmosphérique. Pour les riverains de l'aéroport de Roissy, c'est la double peine. Les 500 000 vols qui ont lieu chaque année, dont une partie se fait de nuit, perturbent leur sommeil. Derrière ce chiffre, il y a une réalité sanitaire. C'est l'accroissement considérable du risque de développer des maladies cardio-vasculaires, synonyme d'une réduction de l'espérance de vie pour les populations qui résident à proximité des aéroports. Et il ne s'agit pas ici d'un problème dont le règlement pourrait se limiter à quelques aménagements superficiels, car c'est aussi un enjeu climatique.

pour que la France atteigne ses objectifs climatiques. L'instauration d'un couvre-feu nocturne de vingt-deux heures à six heures et le plafonnement à 440 000 du nombre de vols annuels à Roissy vous ont été demandés dans un courrier signé

un développement vertueux de l'activité aérienne suppose de pouvoir discuter sans entrave aussi bien de l'apport d'un aéroport que des nuisances qu'il engendre pour les populations locales. Ce constat est précisément à l'origine du concept d'approche équilibrée, défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale et traduit dans le droit européen directement applicable en France. Cette approche privilégie l'appel à trois « piliers » ou leviers d'action pour limiter les nuisances sonores aériennes. En cas de problème de bruit résiduel, le recours à des restrictions d'exploitation peut ensuite être envisagé. Les prévisions de trafic que vous évoquez sont celles qui ont servi à l'établissement des cartes stratégiques de bruit, les CSB. Elles ne revêtent pas de caractère contraignant et ne doivent pas être lues comme des objectifs de développement de trafic. Elles ont été retenues dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire, peu favorable à la conduite d'une réflexion sur les perspectives de développement de l'aéroport, et pour un exercice spécifique, à savoir l'établissement des CSB et du plan d'action qui en découle, Ce plan porte notamment sur des mesures de réduction du bruit relevant des trois premiers piliers de l'approche équilibrée, qui permet, le cas échéant, d'identifier si un problème de bruit subsiste. De fait, le PPBE de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle identifie un problème de bruit résiduel et prévoit le lancement d'une étude d'impact selon l'approche équilibrée. C'est dans le cadre de cet exercice que se fera l'analyse des mesures de restrictions envisagées et de leurs effets sur les nuisances sonores et l'activité économique. La désignation, par le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires, d'une nouvelle autorité compétente permet enfin de s'engager dans cette voie. Le dialogue autour du développement de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et des prévisions de trafic de long terme aura lieu dans ce contexte. La parole

Madame la secrétaire d'État, j'aimerais appeler votre attention sur les projets de rénovation urbaine de la ville de Petit-Quevilly, qui, malgré une candidature particulièrement solide, ne fait pas partie de la liste des communes retenues dans le dispositif des « quartiers résilients commune est engagée dans un projet pour le quartier de la Piscine, qui fait l'objet d'une inscription au titre des quartiers d'intérêt national. La municipalité, avec l'appui de ses différents partenaires, développe un programme d'investissement de plus de 85 millions d'euros. Pour l'heure, malgré des coûts élevés et des difficultés de financement, la commune tient le calendrier initial du projet. Elle a réaffirmé la priorité de ces investissements dans le cadre de son budget pour 2023 et de son programme pluriannuel d'investissement. Parmi les indicateurs quantitatifs de vulnérabilité dévoilés, la ville de Petit-Quevilly, en particulier le quartier de la Piscine, est fortement concernée par plusieurs items des difficultés économiques, sociales et culturelles.

Face à ces enjeux, la municipalité est pleinement investie au travers de projets concrets. Elle s'est engagée dans une politique de transition écologique ambitieuse, avec la création à proximité du quartier de la Piscine d'une forêt urbaine ou encore le projet d'autoconsommation collective et de raccordement à la chaufferie urbaine. national de renouvellement urbain), la ville de Petit-Quevilly a eu à coeur d'être exemplaire et de travailler au-delà de la simple question du bâti et de l'aménagement urbain. Elle a choisi de mettre l'éducation et le sport au centre de son programme, en rénovant par exemple l'ensemble des écoles et le théâtre du quartier. Cependant, la commune a besoin de moyens supplémentaires. Le soutien de l'État au travers du programme « quartiers résilients » lui est donc indispensable, afin qu'elle réussisse la transition du quartier. Ainsi, madame la secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir m'indiquer dans quelles mesures la commune du Petit-Quevilly pourra obtenir les bénéfices de ce classement et de ces crédits.

La démarche « quartiers résilients » vise à s'assurer que la mise en oeuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain, intègre pleinement les enjeux de la résilience, notamment au regard du changement climatique. Un accompagnement et des formations sont ainsi proposés à chaque porteur de projet et les partenaires des « quartiers résilients » apportent leur expertise dans ce cadre. M. le ministre souligne que l'objectif de la résilience sera mis à l'agenda de toutes les revues de projet, dont le format sera adapté, afin d'identifier les marges d'amélioration et de s'assurer que chaque opération contractualisée prenne bien en compte les enjeux de la résilience. Par ailleurs, une cinquantaine de quartiers qui présentent les signes de vulnérabilité les plus marqués pourront bénéficier d'un accompagnement renforcé et de crédits du fonds résilience porté par l'ANRU, complétés éventuellement par des soutiens financiers d'autres acteurs, selon la nature des opérations projetées. Dans ce cadre, une première liste de vingt-cinq quartiers a été récemment retenue, et une seconde le sera à l'automne. Le projet de renouvellement urbain de la commune de Petit-Quevilly présente un bon niveau d'avancement. Il s'agit prioritairement de poursuivre sa mise en oeuvre, afin de respecter les délais d'engagement pour les opérations du NPNRU, soit au plus tard un dépôt des demandes mi-2026, afin que les dotations octroyées octroyées soient pleinement mobilisées et produisent leur effet. Dans cette optique, les services de l'État accompagnent actuellement la commune de Petit-Quevilly sur la dépollution des sols du quartier en vue d'une mobilisation de l'Ademe dans le cadre du fonds vert. La parole

Par manque de temps, je n'insisterai pas sur le fait que les résultats des diagnostics peuvent différer d'un professionnel à l'autre, pas plus que je ne mentionnerai le coût des travaux ou les difficultés pour obtenir, dans certains cas, l'accord des copropriétés. Je me contenterai ce matin d'évoquer la question des petites surfaces. Il n'est pas admissible, madame la secrétaire d'État, qu'à isolation égale, la classification d'un bien diffère sensiblement selon sa taille. C'est pourtant le cas puisque les petits logements ont des surfaces dites déperditives- essentiellement les murs les murs - importantes par rapport à la surface habitable. Ainsi, selon l'Observatoire national de la rénovation énergétique, 63 % des petites surfaces seraient classées E, F ou G, contre 39 % pour l'ensemble du parc. Dans certains cas, les travaux préconisés sont non seulement onéreux, mais aussi et surtout techniquement irréalisables. Que faire quand la seule proposition d'un diagnostiqueur est la pose d'une pompe à chaleur au troisième étage d'un studio en centre-ville ? C'est tout simplement impossible pour des questions d'urbanisme, d'esthétique et de nuisances notamment sonores ... Ma question est très simple : que comptez-vous faire pour remédier à cette situation qui aggrave une crise du logement déjà problématique ? Ne faudrait-il pas donner suite à la proposition de la fédération des diagnostiqueurs, qui préconise la mise en place de coefficients de pondération ? La parole

visant, notamment, les passoires énergétiques : gel des loyers, interdiction de mise en location selon un calendrier progressif, obligation d'audit énergétique lors de la vente. À partir de 2024, certaines aides à la rénovation énergétique seront de manière plus systématique associées à une mesure initiale de la performance du logement par un DPE. La réforme du DPE de 2021 a permis de le fiabiliser. Désormais, le DPE s'appuie uniquement sur les caractéristiques physiques du logement. Il ne recourt qu'à des données d'entrée disposant de justificatifs. Cette refonte apportant plus de fiabilité méthodologique a été accompagnée dès l'été 2022 par une feuille de route ministérielle visant, notamment, à améliorer la qualité de réalisation des DPE. Un arrêté sera publié l'été prochain pour renforcer les obligations de formation des diagnostiqueurs à partir de 2024, ainsi que les contrôles qui s'exercent sur eux. Les recommandations de travaux incluses dans le DPE peuvent être complétées par la réalisation d'un audit énergétique, obligatoire depuis le 1 avril dernier pour la vente de logements classés F ou G en monopropriété, dont les scénarios de travaux sont détaillés et tiennent compte des spécificités du bâti afin d'atteindre la classe B. S'agissant des logements soumis des contraintes architecturales et patrimoniales, leur spécificité est reconnue. Bien évidemment, certains travaux ne pourront être réalisés. Leur performance énergétique peut néanmoins, dans la plupart des cas, être fortement améliorée. La parole est à M. Hervé Maurey, pour la réplique.

que nécessite pour certains territoires une gestion assumée de cette compétence, le législateur, à l'article 1530 du code général des impôts, a ouvert aux EPCI la possibilité de disposer d'une ressource financière fléchée, appelée taxe Gemapi ou aquataxe. La taxe Gemapi fait partie de la liste des taxes spéciales d'équipement (TSE). Ces dernières sont prélevées sur les entreprises et les propriétaires. Si la collectivité choisit de l'instaurer, la taxe vient ainsi s'ajouter aux taxes locales. Son assiette se répartit alors entre la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, mais aussi la cotisation foncière des entreprises. Le taux d'imposition de la taxe Gemapi, appliqué sur chacune de ces taxes, est défini à partir des recettes fiscales de ces de ces dernières en année . La taxe d'habitation étant totalement supprimée à compter de 2023, le poids de la taxe Gemapi, dont l'EPCI- il convient de le préciser -ne vote que le volume du produit et non les taux, ne reposera à partir de l'année 2024 que sur les seuls propriétaires. Cette situation est particulièrement inique, puisque l'objet même de cette taxe est de financer les investissements visant à protéger les personnes et leurs biens, c'est-à-dire toutes les personnes, qu'elles soient propriétaires ou locataires, et tous leurs biens, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers. Madame secrétaire

qui exercent la compétence Gemapi. Le produit de la taxe est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire de l'EPCI. Ainsi, la taxe n'est pas uniquement supportée par les propriétaires, mais elle est également supportée par les contribuables redevables de la CFE et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Les entreprises contribuent donc au paiement de cet impôt. Par ailleurs, l'État a déjà compensé les différentes réformes fiscales pour éviter que la répartition issue de ces réformes ne soit supportée par les contribuables. Enfin, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui prévoit la récupération des charges locatives, serait difficilement applicable à la Gemapi. En effet, cet article permet au bailleur d'exiger le remboursement des dépenses exposées en contrepartie des services rendus liés à l'usage du logement, des dépenses d'entretien courant, des menues réparations et des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement. La Gemapi ne se rattacherait à aucune de ces catégories de dépenses et une disposition spécifique devrait prévoir sa récupération, ce qui risquerait d'ouvrir le champ à des demandes reconventionnelles. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas la possibilité d'une récupération, par le propriétaire, de cette taxe auprès du locataire. La parole

de la cohésion des territoires. Le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre l'engagement de la Première ministre relatif au fonds vert, dispositif inédit visant à accélérer la transition écologique dans les territoires. Je ne peux que saluer cet effort qui s'élève à 2 milliards d'euros. Pour autant, je me permets d'émettre des réserves quant aux modalités de répartition de ce fonds. Je rappelle que les clés de répartition retenues sont la démographie et les besoins de chaque territoire. Arrêtons-nous un instant sur ces deux critères. Envisageons d'abord les besoins. Personne ne peut ignorer les enjeux guyanais en matière de transition écologique. L'urgence est omniprésente. J'en veux pour preuve le nombre important de dossiers déposés auprès de la préfecture. Les demandes ont largement dépassé l'enveloppe de 9 millions d'euros allouée à la Guyane. Parlons maintenant de l'autre critère : la démographie. Dans son ensemble, la classe politique guyanaise est convaincue que les chiffres du recensement sont insincères. Pourtant, ces mêmes chiffres sont employés pour calculer la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités et, dans le cas particulier qui nous concerne aujourd'hui, le fonds vert. Il y a ce sentiment d'injustice qui perdure. La Guyane, on sait très bien la citer et la situer quand il s'agit d'évoquer la richesse de sa biodiversité. une fois de plus, parmi les territoires les moins bien dotés. Bien que ce fonds vert soit globalement fongible avec d'autres aides, mon territoire ne sera jamais suffisamment avantagé pour faire face aux aux enjeux liés à l'accélération de la transition écologique. Je peux vous assurer que ma volonté n'est nullement d'exiger que Pierre soit déshabillé au profit de Paul. Mais il serait opportun que d'autres critères,

Le fonds vert, annoncé en août 2022 par la Première ministre, a pour ambition d'accompagner les collectivités dans leurs projets en lien avec la transition écologique des territoires. Il est doté de 2 milliards d'euros et répond à un triple objectif renforcer la performance environnementale, adapter les territoires au changement climatique, améliorer le cadre de vie. Le déploiement du fonds vert repose sur une répartition des crédits entre régions afin de répondre enjeux spécifiques des territoires. La Guyane a en effet reçu une enveloppe de 9 millions d'euros, qui permettra de mettre en oeuvre divers projets au service de la transition écologique. Comme dans la plupart des autres régions, l'aide demandée au titre du fonds vert excède l'enveloppe déléguée. Ce constat reflète la forte demande des collectivités et leur volonté de participer à l'effort collectif qu'exige la transition écologique. Si la demande de financement globale à l'échelon national se situe à hauteur de 24 % du montant total des projets, les territoires ultramarins observent les taux de financement les plus élevés.

7 dossiers ont été acceptés en Guyane sur la plateforme « Démarches simplifiées » pour un total de 2 millions d'euros de subventions attribuées. Ces projets concernent la prévention des risques d'inondation, l'adaptation au recul du trait de côte ou le tri et la valorisation des biodéchets. L'exercice 2023 a constitué la première année du déploiement du fonds vert, et l'intégralité des crédits devrait être engagée d'ici à la fin de l'année pour soutenir un grand nombre de projets, en métropole et dans les territoires ultramarins. La Première ministre a annoncé

et des outre-mer. Monsieur le ministre, le 3 mai dernier, en vue de la Coupe du monde de rugby, la préfète du Rhône publiait un arrêté visant à expulser les camionnettes dans lesquelles des femmes exercent une activité prostitutionnelle dans le VII arrondissement de Lyon. Initialement circonscrit aux abords du stade lors des pourparlers, le périmètre a été élargi à tout l'arrondissement et concerne désormais des centaines de personnes qui se retrouvent dans une extrême précarité, malgré les tentatives de négociation et les propositions de solutions Pour la majorité de ces femmes, il s'agit non pas de simples camionnettes, mais de leur logement. Dans la journée, elles y dorment, car elles travaillent de nuit. Une mise en fourrière de ces véhicules, outre son coût important, signifie une mise à la rue sans aucune solution d'hébergement alternative. Du fait des multiples expulsions, les associations se trouvent entravées dans leur action pour l'accès aux soins de ces personnes et elles comptent déjà de nombreuses sorties de parcours de soins. Ces expulsions éloignent les personnes des associations, accroissent leurs vulnérabilités et leur insécurité, et les exposent à plus de violences et de risques. La santé des femmes et leur sécurité étant ainsi en jeu, ma question est double. Quelles solutions existe-t-il pour la sécurité de ces personnes si elles se retrouvent soudainement sans camions et donc sans domicile ? Pouvez-vous, monsieur le ministre, suspendre cet arrêté préfectoral afin que de nouvelles négociations avec les parties prenantes s'engagent pour garantir, « en même temps », la tranquillité des riverains et le bon déroulement de la Coupe du monde, tout en protégeant la sécurité et les conditions de vie des personnes concernées, sans rupture du lien avec les

Les abords du stade sont touchés, depuis plusieurs mois, par l'augmentation des faits de violences, notamment à l'encontre des personnes se livrant à la prostitution. Face à ces troubles, un arrêté municipal réglementant le stationnement sur certaines portions et voies du quartier de Gerland a été pris, sans succès. Dans ce contexte, et en vue du public attendu dans les semaines et mois à venir, l'autorité préfectorale était fondée à prévenir ces troubles graves à l'ordre public dans un périmètre restreint, soit dans une vingtaine de rues seulement autour du stade de Gerland, et non sur l'ensemble de l'arrondissement. La mise en oeuvre de cet arrêté, qui se borne à interdire le stationnement des véhicules dans lesquels s'exerce une activité de prostitution, n'a pas pour vocation d'expulser ces femmes ni de saisir leurs véhicules ; il leur appartient seulement de respecter l'arrêté et de ne pas stationner dans le périmètre interdit.

La commission départementale de lutte contre la prostitution et le proxénétisme, instituée en 2016 et exerçant auprès du préfet de département, met en oeuvre la prévention et l'accompagnement de ce public. C'est sa mission prioritaire. Des résultats ont Des résultats ont d'ores et déjà été obtenus dans le département du Rhône : sur un total de 52 dossiers suivis entre décembre 2018 et septembre 2022, avec l'appui de deux associations agréées par l'État- l'Amicale du Nid

des outre-mer. Monsieur le ministre, l'immigration clandestine est incontrôlée. L'État n'arrive pas à juguler cette pression illégale. Mon département des Alpes-Maritimes, que représente aussi la sénatrice Patricia Demas, en est tout un symbole : 40 000 migrants clandestins ont été interpellés sur toute l'année 2022 à la frontière italienne, selon le préfet. Cette défaillance ne se limite pas seulement à une absence de contrôle, elle porte également sur l'explosion du nombre de jeunes clandestins, dits mineurs non accompagnés Le président du département, les parlementaires, les maires ne cessent de lancer un cri d'alarme face à cette accélération inquiétante. Plus de 5 000 de ces mineurs sont entrés dans notre pays, dont 2 000 dans les seules Alpes-Maritimes. Les structures sont débordées par cette saturation qui dépasse largement la mission de protection de l'enfance, malgré des efforts importants du département de l'ordre de 20 millions d'euros. Je peux en témoigner, puisque j'ai été président du foyer de l'enfance. Symbole supplémentaire de cette embolie, le préfet des Alpes-Maritimes ne cesse de prendre des arrêtés de réquisition à répétition d'équipements tantôt privés, comme un hôtel à Antibes, à Châteauneuf-de-Grasse ou encore à Biot, tantôt publics, comme un gymnase à Menton. Ces réquisitions sont réalisées à marche forcée, sans aucune concertation ni aucun échange avec les maires, qui sont clairement mis devant le fait accompli. L'État ne peut multiplier ces réquisitions et faire peser sur les maires le poids de ses propres carences sur les territoires. Au-delà du fait qu'il devrait revenir à l'État d'assumer pleinement cet accueil,

Le parquet de Nice a également mobilisé des ressources nouvelles afin d'accélérer la prise des ordonnances de placement de façon à réorienter des mineurs vers d'autres départements.

a réquisitionné deux structures afin de permettre la prise en charge des mineurs. Une résidence hôtelière d'Antibes a ainsi été mise à disposition pendant un mois en mars et un gymnase a été mobilisé à Menton pendant huit jours en avril. jours en avril. Dans les deux cas, les maires des communes concernées ont été préalablement informés par le préfet des raisons pour lesquelles ces réquisitions avaient dû être prises, à la demande du conseil départemental. La coopération entre le conseil départemental, le préfet et les maires me semble de bon aloi. Elle fonctionne correctement. Nous recherchons activement aujourd'hui toutes les solutions utiles à l'exercice par la collectivité départementale de la mission d'aide sociale à l'enfance

préoccupante de la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. J'ai rédigé ces courriers à la suite de visites de l'établissement. Sa capacité d'accueil est de 85 places alors qu'il compte aujourd'hui 147 détenus, parfois plus, soit un taux d'occupation de plus de 170 % ! Dans un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, rendu public le 18 juillet 2022, le constat est clair : la maison d'arrêt de Saint-Brieuc est l'une des plus surpeuplées de France. Ce même rapport fait état également de l'« indignité » des conditions de détention : infiltrations d'eau, moisissures, trous dans les murs, mobilier détérioré ou manquant, absence d'intimité dans les WC ouverts sur les cellules à trois lits superposés, état d'hygiène déplorable des sols et des lits, manque d'espace pour les gestes du quotidien.

encore plus urgents à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 24 au 25 mai dernier. Il est impératif de garantir une hygiène correcte et de bonnes conditions de restauration pour les détenus, mais aussi pour le personnel. Une rénovation d'ampleur paraît nécessaire, voire une reconstruction sur un autre site, comme l'a souligné le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guihard : « Le territoire briochin est disposé à faire émerger un lieu qui puisse accueillir un nouvel équipement pénitentiaire. » Dans l'attente, une régulation des entrées en lien avec l'autorité judiciaire serait nécessaire pour éviter une surpopulation : quatre détenus dans onze mètres carrés, cela relève de l'indignité ! Les conditions de travail sont donc particulièrement difficiles pour le personnel de surveillance. Monsieur le ministre, quel est votre projet pour la maison d'arrêt de Saint-Brieuc en termes immobilier et, dans l'attente, pour réguler les entrées et assurer un accueil digne ? La

le projet que porte mon collègue garde des sceaux pour une meilleure efficacité de la réponse pénale, de meilleures conditions de travail pour les agents pénitentiaires et des conditions de détention plus

La construction d'un centre pénitentiaire à Vannes dans le cadre de ce programme permettra une meilleure prise en charge de la population pénale au sein de ces territoires. En outre, les services de l'administration pénitentiaire ont bien conscience des conditions de détention à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. La direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes met tout en oeuvre, croyez-le, pour désencombrer l'établissement, notamment en orientant les personnes détenues vers d'autres établissements pénitentiaires moins surpeuplés. Par ailleurs, les services de l'administration pénitentiaire travaillent étroitement avec le parquet près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de remédier à la situation de cette structure. Les chiffres sont un peu plus impressionnants que ceux que vous citez, puisque, au 1 juin 2023, le taux d'occupation de la structure était de 193 %, soit 164 personnes détenues pour 85 places.

de solution à court terme. Cette modalité d'exécution des peines, qui permet aux personnes détenues en toute fin de peine de bénéficier d'un contrôle accru ainsi que d'une prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en milieu ouvert, est pleinement mise en oeuvre par l'autorité judiciaire dans cet établissement

alertés par le barreau de Marseille et les représentants du monde économique sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir ce projet s'il voyait le jour. Une étude d'impact a été menée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille. La conclusion est sans appel les acteurs du monde du droit font vivre tout un secteur qui se videra de sa substance si les juridictions sont délocalisées en périphérie du coeur de la cité phocéenne.

De surcroît, sept avocats sur dix sont localisés à moins de dix minutes à pied du palais de justice. Si la cité judiciaire sort de l'hypercentre, la plupart des professionnels du droit vont devoir transférer leur activité et leur cabinet. Ma question est simple : pourquoi délocaliser l'ensemble

Trois options sont envisagées pour la construction d'une cité judiciaire : sur un site en centre-ville pour 450 millions d'euros et six ans de construction, sous réserve de la faisabilité technique un terrain à la Capelette, sous réserve de difficultés dues à la proximité d'un centre de traitement des déchets ; sur un terrain à Euroméditerranée

ans ou construire un simple palais de justice sur ce terrain, le conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce restant à Monthyon pour un budget total de 370 millions d'euros et quatre ans de construction. Il ne s'agira alors plus d'une cité judiciaire.

La Chancellerie propose dans ce dernier cas d'utiliser le site du palais Monthyon pour l'école du barreau et une annexe de l'École nationale de la magistrature. Il ne s'agit pas d'abandonner le bâtiment. Les textes défendus par le garde des sceaux actuellement devant le Parlement un plan d'embauche historique de magistrats, de greffiers et d'attachés de justice. Ils pourraient être formés à Marseille. Nous ne méconnaissons pas l'enjeu symbolique et, surtout, économique que constitue une implantation judiciaire. C'est pourquoi le garde des sceaux a souhaité que cette réflexion se poursuive et puisse s'articuler autour d'autres enjeux locaux. La concertation engagée par le préfet est la seule qui permettra d'identifier la solution la plus adaptée et, ainsi, d'éclairer la décision du Gouvernement. La

est au coeur de la cité, où elle doit se redresser fièrement pour incarner l'État et l'autorité. La parole est à M. Ronan Le Gleut, étrangères. Monsieur le ministre, par arrêté du 30 novembre 2020, un dispositif de recueil et de traitement des signalements de faits de harcèlement, de discrimination ou d'agissements sexistes ou violents a été mis en place au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, avec la création d'une cellule encadrée par un « référent écoute ». Des présomptions de faits de cette nature existent dans divers consulats, notamment au Canada, et entraînent de lourdes conséquences, tant pour les agents du ministère que pour la France et les Français de l'étranger dysfonctionnements dans ces consulats ont pour corollaires des difficultés dans le service rendu aux Français de l'étranger et l'image de la France est ternie dans les médias étrangers. En mars dernier, l'Assemblée des Français de l'étranger a souhaité, comme elle l'avait fait l'année précédente, entendre en audition le référent écoute, mais le ministère l'a refusé, alors que ce sujet concerne pourtant les Français de l'étranger. Je souhaite donc connaître des statistiques précises sur le sujet : nombre de signalements, nombre d'enquêtes diligentées ainsi que nombre et nature des décisions prises à la suite de ces signalements, notamment pour les agents ayant dénoncé ces faits.

Dans 98 % des affaires pour lesquelles la direction des ressources humaines a été saisie, une action a été menée, les 2 % restants étant classés, car ils ne relevaient pas d'un harcèlement, d'un agissement sexiste ou d'une discrimination. Pour les cas les plus graves, des enquêtes sont diligentées, qui sont menées avec beaucoup de rigueur et de façon indépendante. Le principe est simple : tolérance zéro. Lorsque l'enquête met en lumière des comportements inappropriés ou des faits de harcèlement,

à une certaine prudence avant de vous prononcer sur une affaire sur la simple foi d'articles de presse, qui ne donnent à lire qu'une version des faits. Ces situations sont rarement simples et les responsabilités sont parfois partagées. Il faut du temps pour aller au bout d'un dossier, c'est un gage de rigueur, d'objectivité et de justice. Croyez-le bien, aucune affaire n'est abandonnée.

Cela me rappelle un autre cas emblématique, celui de la circulaire relative aux relations entre nos postes diplomatiques et les conseillers des Français de l'étranger, que le ministère refuse de nous communiquer, alors que celle qui avait été écrite sur le même sujet, lorsque Philippe Douste-Blazy était ministre, était publique. Il est temps de lever le grand secret qui règne depuis quelques années au sein de ce ministère pour mettre fin à des situations disparates et parfois inacceptables. Le Parlement joue un rôle essentiel dans la bonne marche démocratique de notre pays en assurant le contrôle de l'action gouvernementale ... Veuillez conclure, mon cher collègue. ... et nous allons réfléchir aux moyens que nous offre le règlement du Sénat pour accéder aux informations que le ministère de l'Europe et des affaires étrangères nous refuse. à Mme la ministre de la culture. Monsieur le ministre, je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur les obligations de fouilles archéologiques préventives qui s'appliquent aux opérations d'aménagement. La loi impose aux collectivités la réalisation de fouilles lorsque leurs projets d'aménagement ou de construction sont susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Force est de constater que la mise en oeuvre de cette obligation pose des difficultés dans bon nombre de territoires ruraux. Dans le département dont je suis élu, l'Allier, la situation de la communauté de communes de Lapalisse illustre bien ce phénomène : un projet d'extension d'une zone d'activités économiques est à l'étude, pour un montant de 1,3 million

Les collectivités sont dans l'incapacité de supporter de telles dépenses ou sont contraintes de le faire au moyen de montages financiers doublant le prix de vente du mètre carré aménagé, bien loin des prix moyens pratiqués sur le territoire ... Ce cas n'est pas isolé ! Des situations similaires ont été vécues à Dompierre-sur-Besbre et à Varennes-sur-Allier, qui ont dû renoncer à leur projet devant le coût exorbitant des fouilles, et des difficultés ont été rencontrées à Gannat et à Creuzier-le-Neuf.

des travaux. Il convient que l'État prenne conscience de cette difficulté et apporte des solutions pour mieux accompagner le développement en ruralité, qui risque par ailleurs d'être encore plus contraint avec l'application du «

Afin d'anticiper les enjeux archéologiques de leurs projets et de réduire le coût des fouilles, les communes peuvent interroger en amont les Drac pour connaître la sensibilité archéologique des terrains considérés. Le financement des fouilles repose essentiellement sur les maîtres d'ouvrage,

Pour les prises en charge, les communes situées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement peuvent donner mandat à l'opérateur de fouilles pour encaisser directement l'aide accordée, ce qui permet d'éviter une sortie de trésorerie. Par ailleurs, l'impact du coût de la fouille sur l'équilibre financier du projet fait partie des critères d'éligibilité de la subvention. En moyenne annuelle, entre 2016 et 2022, 44 % des fouilles ont reçu annuellement un soutien financier de l'État

le diagnostic a révélé une forte densité de vestiges archéologiques, dont la chronologie s'étire du second âge du fer au Moyen Âge central. Après échange avec les collectivités- voici la mesure qui va vous intéresser -, il a été convenu que l'emprise globale de la fouille serait scindée en trois

à Mme la ministre de la culture. Dans une région à forte identité comme la Corse, la culture, l'histoire, le patrimoine, sont des marqueurs importants, qui unissent le passé au présent pour mieux se projeter dans l'avenir. Depuis plusieurs années, sous l'impulsion des anciens départements et de la collectivité de Corse, avec le concours des services de l'État, mais aussi de l'Union européenne, notre île a développé une politique culturelle proactive, qui s'est notamment traduite par la création de musées témoignant de l'histoire insulaire, une mise en valeur qui constitue aussi un vecteur d'attractivité touristique qu'il convient de consolider. Il se trouve que la Corse, en raison de sa position centrale en Méditerranée occidentale, a longtemps été un carrefour ; les fouilles archéologiques attestent de cette richesse historique. Avant qu'elle ne dispose des infrastructures d'accueil adéquates, des objets découverts sur le territoire insulaire ont été transportés ailleurs et ne sont pas exposés dans les musées de l'île. Certains datent du néolithique, d'autres de l'âge du bronze, beaucoup du Moyen Âge. quelques exemples notables, comme la statuette datant du néolithique dite Vénus de Campu Fiureddu, découverte au début du XX siècle à Grossa, près de Sartène, et qui est exposée au à Londres, alors qu'elle pourrait l'être à Sartène

L'intercession fructueuse de la ministre de la culture en faveur du retour en Corse de la le mois dernier a pu se faire parce qu'il y avait une vente aux enchères en cours. Néanmoins, bon nombre des oeuvres qui pourraient être conservées en Corse appartiennent à des musées situés à l'étranger. ma demande consiste à vous solliciter pour savoir comment nous pourrions procéder pour les rapatrier dans des musées insulaires, qui restent les meilleures vitrines de l'histoire de la Corse. Si vous souscrivez à ce projet, sachez que ce travail risque d'être long et sinueux, dans un environnement juridique impliquant des législations nationales différentes.

leur situation actuelle semble peu contestable en droit et seule la négociation de prêts pourrait être entreprise pour permettre leur présentation en Corse. Bien que le ministère de la culture soit évidemment sensible à la protection du patrimoine en général, y compris

qu'elles soient originaires de Corse ou d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ma collègue ministre de la culture reste très attentive au sort de la et à la possibilité qu'elle retourne en Corse, qui reste évidemment sa destination privilégiée. Elle s'est entretenue à ce sujet avec le président du conseil exécutif de la Corse. Les services du ministère, en administration centrale et en Drac, sont pleinement mobilisés auprès de la collectivité de Corse et de la commune de Brando

préalablement concernés. Si ce dispositif est très attendu, certaines communes nouvellement entrantes perdront le bénéfice de la taxe d'habitation sur les logements vacants, lorsqu'elles l'avaient instituée. Quand une commune perçoit cette taxe, cela sous-entend que la fiscalité ne produit pas les effets

Demain, l'objectif « zéro artificialisation nette » freinera le développement des villes et les contraintes énergétiques pour la location accentueront les problèmes que des dispositifs fiscaux ne sauront seuls résoudre.

Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui revient sur une réforme importante de la loi de finances pour 2023. Comme vous le relevez, une solution était vivement attendue pour répondre aux difficultés liées à l'attrition du nombre de logements disponibles dans certaines communes, notamment touristiques. C'est à cette fin que le Parlement a prévu, dans la loi de finances pour 2023, l'extension du zonage de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) et de la majoration facultative de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) au-delà des seules communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Cette extension vise notamment des communes touristiques qui, sans atteindre ce seuil de population, sont confrontées à une forte tension immobilière, par exemple en raison d'une proportion élevée de résidences secondaires. Après une phase de consultation, le décret procédant à la modification de la liste des communes concernées devrait être très prochainement publié. L'entrée dans le nouveau zonage se traduira par l'assujettissement à la TLV des logements vacants, y compris pour les logements situés sur le territoire de communes qui avaient préalablement institué la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV). L'incitation à faire cesser la situation de vacance de ces logements sera ainsi accrue, en les imposant dès la première année de vacance à un taux national, relevé dans la loi de finances pour 2023 et qui est, en moyenne, plus élevé que celui de la THLV.

Les promesses n'engagent que ceux qui y croient et l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité s'est insurgée contre le fait que, dans certaines collectivités, le montant de la compensation théorique était nettement inférieur au montant de CVAE qui aurait été perçue en 2023.

Vous le savez, il a été institué par la loi de finances pour 2023 un fonds vert ayant pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la lutte contre la crise climatique et contre l'effondrement de la biodiversité.

relative au déploiement du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires demande ainsi aux préfets de s'assurer que les collectivités concernées par la suppression de la CVAE « bénéficient [ ...] du fonds [ ...] à hauteur de la compensation prévue Or, s'il était bien convenu que les collectivités bénéficieraient d'un accès favorisé au fonds vert pour retrouver une compensation intégrale de la CVAE, intégrer de cette manière la compensation au sein du fonds vert est de nature à rendre plus difficile l'accès au fonds lui-même pour les collectivités bénéficiant de la compensation.

En matière énergétique, le Gouvernement a protégé les collectivités locales, notamment avec le bouclier tarifaire, qui a limité pour les petites collectivités la hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité, et avec l'amortisseur électricité pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier. Au-delà de ce soutien spécifique, le bloc communal bénéficie en 2023 Au-delà de ce soutien spécifique, le bloc communal bénéficie en 2023 d'une revalorisation forfaitaire des bases d'imposition de 7 %. Les recettes fiscales des collectivités devraient ainsi rester dynamiques en 2023, notamment avec la hausse du produit de la TVA, évaluée à 5,1 %.

La pompe à chaleur hybride, association d'une pompe à chaleur électrique de puissance optimisée à une chaudière gaz à très haute performance énergétique, permet de diminuer la consommation de gaz chez les particuliers et de préserver l'équilibre du système électrique en hiver. Face aux risques pesant sur la sécurité d'approvisionnement, pourquoi se priver d'un tel outil de flexibilité ? L'interdiction des chaudières au gaz aurait également des effets dévastateurs sur la pointe électrique et la sécurité d'approvisionnement. Les écarts entre offre et demande pourraient, s'ils se cumulaient, atteindre lors des pointes lors des pointes hivernales en 2050 entre 30 et 50 gigawatts, voire davantage si les interconnexions avec les pays voisins n'étaient pas mobilisables ou si des solutions de flexibilité plurijournalières et saisonnières ne permettaient pas de compenser l'intermittence de la production des Aucun scénario de RTE n'anticipe une telle situation. De plus, l'interdiction des chaudières au gaz exigerait des investissements supplémentaires sur le réseau électrique, alors que les investissements nécessaires sur le système électrique à l'horizon de 2050 sont déjà estimés entre 750 milliards En revanche, le développement des gaz verts ne nécessite pas d'investissements lourds : l'investissement nécessaire sur les moyens de production et les infrastructures est évalué à 150 milliards d'euros. Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur l'interdiction d'installer des chaudières au gaz dans les logements et savoir

le ministre délégué. Monsieur le sénateur Longeot, je vous remercie de votre question. Vous le savez, l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, fixé par le Président de la République, représente un défi immense et passera avant tout par la décarbonation des grands secteurs, comme celui du bâtiment. L'enjeu est d'utiliser toutes les solutions décarbonées- il n'y a pas de formule magique -dans les bâtiments qui ne dépendent pas d'énergies massivement importées, comme le gaz. C'est un enjeu de souveraineté pour notre pays et cela permettra dans le même temps de garantir plus de confort et des baisses de facture pour les Français. Le Gouvernement

La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui m'a chargé de répondre à votre question, a insisté sur la nécessité d'une sortie progressive et respectant plusieurs principes. D'abord, il disposer de solutions de substitution décarbonées. Ces solutions existent, elles sont compétitives et elles sont de plus en plus produites en France ; je pense aux pompes à chaleur, aux réseaux de chaleur, au solaire ou encore à la géothermie. prendre en compte les contraintes techniques locales, notamment l'impact sur le réseau électrique et sur notre système énergétique, comme vous l'avez souligné. Enfin, il faut associer les acteurs de la filière. Ma collègue a annoncé récemment le lancement d'une concertation publique sur la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage. J'engage toutes les parties prenantes à y contribuer.

Parcoursup a imposé la généralisation de la sélection aléatoire et il crée un stress pour les élèves, qui doivent arrêter des choix de spécialité engageant leur avenir dès la seconde ; les élèves des filières technologiques et professionnelles en sont les premières victimes. En réalité, beaucoup de bacheliers arrivent en septembre dans une filière où ils ne sont pas à leur place, ce qui les conduit à l'échec scolaire. Dans un rapport publié en 2020, la Cour des comptes soulignait l'opacité de certains critères de sélection

Je vous propose d'abord d'écouter les lycéens, au travers des données issues d'une étude d'Ipsos rendue publique en septembre 2022. Plus de la moitié- 58 % -des lycéens interrogés

Nous avons donc amélioré la transparence de Parcoursup, apporté des informations plus claires sur les critères d'examen des voeux par les commissions d'enseignants- non, Parcoursup n'est pas un « algorithme », ce sont bien des enseignants qui examinent les dossiers -et nous renforçons dès cette année l'efficacité de la phase principale pour apporter des réponses plus vite et réduire le sentiment d'attente. Ce processus d'amélioration se poursuivra. C'est également le cas pour les Ifsi. Le ministre de la santé a lancé une grande concertation avec les professionnels pour engager une réforme de la formation dès la rentrée de 2024.

et de la jeunesse. Madame la ministre, j'ai été sollicité par plusieurs chefs d'établissement d'écoles privées sous contrat d'association, qui dénoncent une dégradation des conditions dans lesquelles ils doivent effectuer leurs missions et dressent un constat alarmant de la situation Le climat général est particulièrement tendu, comme le montrent la hausse des demandes de disponibilités et de congés de formation ainsi que l'augmentation du nombre de démissions et de ruptures conventionnelles. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le malaise ressenti par les enseignants et chefs d'établissement des écoles privées sous contrat : absence de médecine du travail, manque de ressources humaines et matérielles pour bien accompagner les élèves,

avec notamment des différences de salaires incompréhensibles pour des temps de travail pourtant identiques, voire supérieurs. Les candidats sont logiquement de moins en moins nombreux, et les remplacements plus difficiles à pourvoir. Ces enseignants et chefs d'établissement ont la volonté de bien faire leur métier au service des élèves, mais ils estiment que les moyens alloués sont insuffisants et que leurs missions, pourtant essentielles, en pâtissent. Madame la ministre, quelles sont les Madame la ministre, quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à cette situation et pallier les difficultés que rencontrent les écoles privées sous contrat d'association, leurs enseignants et leurs chefs d'établissement ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le

Dans le second degré, il est permis aux maîtres qui souhaitent assurer les fonctions de chef d'établissement de réduire leur service d'enseignement dans des conditions plus favorables que celles de l'ensemble des maîtres, ce qui leur permet de garder un lien avec l'État et de poursuivre leur carrière d'enseignant. Par ailleurs, le versement des forfaits par la puissance publique permet cette prise en charge des personnels d'accompagnement éducatifs ou administratifs. Ces forfaits sont calculés en référence au coût d'un élève de l'enseignement public. Ainsi, la rémunération des chefs d'établissement est intégrée dans le forfait d'externat.

Cette revalorisation vise à harmoniser les grilles de rémunération des agents non titulaires du public et du privé. De plus, ces maîtres bénéficieront d'une partie des mesures de revalorisation transversales qui s'appliqueront à tous les enseignants : revalorisation de l'indemnité de suivi des élèves,

Néanmoins, une définition commune est possible : « Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. » Cette définition est issue de l'avis du Conseil économique et social du 24 février 1993. Il existe deux types de bénévolat : informel, lorsque l'on aide

Certes, la Cour de cassation a pu admettre que le travail effectué par un individu en vue de sa propre insertion sociale était susceptible de générer un pécule et des avantages, à condition que ceux-ci ne relèvent pas d'une relation salariée. Cependant, ce dispositif demeure très largement isolé et conduit à une sous-valorisation du bénévolat en France, dans toutes les catégories d'âge, d'activité et de population qui s'y investissent pleinement. Pour récompenser et remercier les milliers de bénévoles de leur aide précieuse et de leur engagement auprès de la population, il serait pourtant possible de leur offrir une gratification, sous quelque forme que ce soit : chèque-vacances, cotisations sociales, valorisation de droits à la retraite, chèque emploi service universel (Cesu) préfinancé. Le désintéressement de nos bénévoles ne justifie aucune ingratitude de notre part. Madame la ministre, quel dispositif le Gouvernement entend-il mettre en place afin de remercier les bénévoles pour tous les services qu'ils rendent au quotidien ?

deux critères principaux : l'absence de rémunération et l'absence de lien de subordination. La notion de contrepartie financière correspond à une rémunération directe- en espèces -, ou indirecte- en nature -, dont la valeur peut être susceptible de caractériser une activité intéressée.

atout indispensable dans la lutte contre l'exclusion et l'isolement des jeunes, en particulier en zone rurale, et cela depuis plus de quarante ans. En Dordogne, département dont je suis élu, les cinq missions locales permettent un maillage efficace du territoire. Cette connaissance du terrain leur permet de saisir les problématiques spécifiques auxquelles chaque jeune est confronté. Leur connaissance du terrain est nourrie, aussi,

etc. Les missions locales sont un acteur de proximité privilégié pour la jeunesse. À l'heure où les services publics désertent de plus en plus nos territoires, elles jouent un rôle majeur en matière de lutte pour l'égalité des chances. Vouloir les coupler à un algorithme d'orientation désincarné est un non-sens. Dématérialiser à l'excès, c'est déshumaniser, créer une barrière, un obstacle supplémentaire, pour des jeunes déjà déconnectés, exclus. Rien ne remplacera l'humain ! Nous devons Nous devons faire confiance aux agents des missions locales, car leur expertise en matière d'accompagnement de notre jeunesse n'est plus à démontrer. Madame la ministre, les usagers, les personnels et les partenaires des missions locales sont inquiets. Quelles garanties comptez-vous leur donner ?

qui proposent un accompagnement de grande qualité aux jeunes en difficulté. Ainsi sont-elles naturellement appelées à jouer un rôle dans le cadre de France Travail,

d'engagement jeune (CEJ). La gestion des outils et des dispositifs d'accompagnement continuera donc d'associer étroitement les missions locales et Pôle emploi. Pour ce qui concerne la gouvernance, France Travail jeunes contribuera pleinement à pleinement à élaborer les feuilles de route annuelles pour le public jeune de chaque territoire, lesquelles comprendront un retour sur les résultats, année par année, ainsi qu'un diagnostic de la situation actuelle, et détailleront les objectifs communs en matière de repérage, d'accompagnement et de retour à l'emploi des jeunes.

entre les missions locales et leurs financeurs. Le conventionnement direct avec l'État et les collectivités est maintenu. De même, les missions France Travail jeunes pourront, à l'instar des missions locales actuellement, prendre l'initiative du pilotage et être garantes de projets directement portés auprès de l'État et des collectivités dans le cadre de la contractualisation. J'y insiste, les missions locales seront étroitement intégrées dans France Travail et continueront d'assumer leurs missions d'accompagnement des jeunes, mais en s'insérant dans un écosystème imbriqué, rationalisé, et en partageant des objectifs communs. La parole est à M. Hervé Gillé, et de l'insertion. Madame la ministre, 607,75 euros, voilà le montant perçu par une personne seule au RSA, ce revenu de solidarité active qui couvre en France 3,85 millions de personnes. Dans le cadre de son plan de refonte de la relation au travail, le Gouvernement envisage de renforcer les mesures contraignantes pour les allocataires du RSA, en conditionnant le versement de ce dernier au suivi de parcours intensifs d'« heures d'activités »- au nombre de quinze Qu'en est-il exactement de cette intention ? Il est essentiel d'évaluer attentivement les risques induits par de telles mesures et de s'assurer que les politiques mises en oeuvre favorisent une réinsertion durable plutôt que des résultats à court terme. Cette nouvelle conditionnalité du versement du RSA est actuellement testée dans plusieurs départements. Les conclusions de ces expérimentations sont attendues afin d'orienter nos futures réflexions sur cette question. Nous espérons que le Gouvernement sera capable de les entendre et d'adapter sa politique. Le RSA est déjà conditionné aux engagements des allocataires par un contrat avec des professionnels accompagnants sur le plan social et professionnel. Pouvez-vous préciser vos orientations ? Voulez-vous renationaliser le RSA ? Le changement d'organigramme de l'organisation du versement du RSA, donc la remise en question de la place des départements dans le cadre de cette réforme, alertent les collectivités. Voulez-vous placer les départements sous tutelle ? Les discussions doivent se poursuivre pour trouver des approches sociales qui soutiennent réellement l'autonomie des allocataires du RSA et répondent aux enjeux socioéconomiques tout en laissant les départements en première ligne, pour garantir une véritable politique de proximité.

Il s'agit d'alimenter la réflexion afin d'améliorer l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Nous avons donc lancé un grand dispositif de parangonnage : cet exercice